Monsieur le président du Sénat a reçu de Mme la Première ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 19 juin 2023 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du lundi 3 juillet 2023. Par ailleurs, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement confirme l'ordre du jour établi de façon prévisionnelle par la conférence des présidents qui s'est réunie mercredi 14 juin dernier. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame, messieurs les rapporteurs,

Elle a trahi sa culture ouvrière, elle a trahi son génie industriel, elle a trahi son attachement au progrès, à l'innovation technologique et à la production manufacturière. Les chiffres sont sans appel : en quarante ans, six cents entreprises fermées, 2,5 millions d'emplois industriels détruits, des territoires laissés à l'abandon, une part de l'industrie dans la richesse nationale tombée de plus de 20 % à un peu plus de 10 % tandis qu'elle restait stable chez nos principaux partenaires européens- l'Allemagne et l'Italie. Avec le Président de la République, nous voulons maintenant ouvrir une nouvelle ère de réindustrialisation nationale et européenne : c'est l'objet des décisions que nous avons prises depuis plus de six ans ; c'est l'objet de ce projet de loi sur l'industrie verte. Nous disposons maintenant d'une base nationale pour engager cette réindustrialisation. En effet, cette majorité a eu le courage de réformer la fiscalité du capital, ce que personne n'avait fait avant nous : il n'y a pas d'industrie sans capital et taxer toujours plus le capital, c'est taxer l'industrie et renoncer à toute ambition industrielle ! Nous avons mis en place des dispositifs pour améliorer la formation

90 000 emplois industriels. Nous disposons aussi d'une base européenne, résultat d'une longue confrontation avec une idéologie européenne dépassée qui refusait systématiquement, contrairement à ce qui se fait en Chine ou aux États-Unis, qu'un État soutienne, par des subventions ou des crédits d'impôt, le développement d'une industrie à ses débuts. Avec le Président de la République, nous avons obtenu cette révolution idéologique consistant à laisser les États membres apporter des soutiens financiers au développement de leur industrie sous forme de subventions ou de crédits d'impôt. Nous avons obtenu cette autre révolution consistant- Dieu sait que cela devrait être de bon sens -à protéger nos technologies

Après la crise de la covid, chacun a compris qu'il fallait réorganiser les chaînes de valeur, arrêter d'être trop dépendants des autres nations pour les approvisionnements essentiels et faire revenir sur notre sol les approvisionnements critiques et les chaînes de valeur stratégiques. Parmi ces circonstances, il en est une des plus difficiles : l'accélération du changement climatique, qui montre qu'il n'y a désormais pas d'autre issue que de prendre le problème à bras-le-corps et d'y apporter des réponses massives, rapides et efficaces. À partir de là, maintenant que nous avons cette base nationale et cette base européenne et que nous faisons face aux circonstances que je viens de décrire, nous avons devant nous des choix politiques qui sont simples et qui doivent être tranchés. Il y a trois choix possibles. Le premier choix, c'est le : on continue comme avant, la croissance pour la croissance, l'ouverture de sites pour l'ouverture de sites, et peu importe le climat le climat ! Ce serait criminel pour la planète, criminel pour les générations futures et, de toute façon, inacceptable pour nos compatriotes. La croissance pour la croissance au détriment du climat est une impasse. deuxième choix, c'est la décroissance. Je sais qu'elle a la faveur de certains en France. Je tiens à dire à quel point elle conduira à la relégation de la nation française,

: nos compatriotes ne vont pas arrêter d'acheter des voitures, des vélos, des batteries ou des pompes à chaleur, mais, au lieu d'acheter des produits fabriqués sur notre territoire avec nos technologies et nos emplois, ils achèteront les mêmes produits importés, réalisés dans des conditions environnementales moins satisfaisantes. Avec la décroissance, nous sommes perdants sur tous les tableaux : celui de l'emploi, celui de la richesse et celui du climat.

verte. Qu'entend-on par industrie verte ? Deux choses distinctes, mais complémentaires. L'industrie verte, c'est d'abord la décarbonation de l'industrie existante : on ne construira pas l'industrie de l'avenir sur les ruines de l'industrie du passé. Tous ceux qui nous ont vendu ces sornettes pendant des années et des décennies comme quoi il fallait faire table rase des vieilles industries pour construire dessus des industries nouvelles se trompaient totalement sur le lent processus qui permet d'améliorer les technologies, de profiter des savoir-faire passés pour construire ceux de l'avenir. L'industrie existante, c'est 18 % des émissions actuelles de CO2 en France. Avec ce projet de loi, nous voulons accélérer la décarbonation des grands sites industriels français.

C'est ce que j'appelle les : les pompes à chaleur, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les batteries électriques et l'hydrogène vert. Ces cinq technologies clés feront la différence entre les nations qui réussissent au XXI siècle et celles qui importent et qui sont dominées.

De ce point de vue, contrairement à ce que j'ai entendu dire parfois, l'industrie verte n'est pas une contradiction dans les termes : c'est une évidence et même une tautologie. Si nous voulons une industrie, elle doit être verte et, pour que nous soyons verts, nous avons besoin de notre industrie. Alors, comment faire pour avancer dans la direction de la croissance verte que nous vous proposons et qui nous paraît la seule option raisonnable pour la nation française ?

D'abord, ce qui compte le plus pour un industriel qui veut investir en France, ce qui est le plus difficile à trouver, ce qui pose le plus de problèmes, c'est le foncier. Il est extraordinairement difficile en France, pour un industriel qui veut investir, d'avoir accès à du foncier présentant les caractéristiques voulues.

il est prêt à l'emploi. » La seconde mesure consiste à rehausser la créance environnementale au rang des créances privilégiées pour récupérer 25 % des sommes nécessaires pour dépolluer les sites. C'est un geste politique fort que de faire remonter ces créances environnementales au rang des créances privilégiées. du « zéro artificialisation nette » (ZAN), ... Ça, on verra ... ... qui a fait couler beaucoup d'encre et ouvert beaucoup de débats parfaitement légitimes. La proposition est de compter à part les projets industriels majeurs, ainsi que tous ceux qui contribuent aux chaînes de valeur du développement durable. Une fois que vous avez votre site et que vous voulez construire votre usine, le deuxième obstacle auquel vous vous heurtez en France, c'est la lenteur des procédures : nous mettons trop de temps à accorder les autorisations. Nous voulons, avec ce projet de loi, diviser par deux

les différentes autorisations administratives. Cela se fera sans affecter les exigences environnementales ni la consultation publique, dont la durée passera d'un mois à trois mois.

L'État prendra la main, de manière à accélérer les procédures, sur ce qui concerne le raccordement électrique, le permis de construire ou encore la modification du plan

Troisième étape de la construction d'une usine, pas la moindre : l'accès à des financements. Pour des usines de batteries électriques, d'hydrogène vert ou d'électrolyse,

Nous avons besoin de financements dans un moment- je crois l'avoir dit clairement hier -où il faut redresser les comptes publics et où, par conséquent, les financements publics sont rares. Nous allons donc mobiliser l'épargne des Français. Nous vous proposons de mettre en place un plan d'épargne avenir climat (Peac) disponible pour tous les mineurs, bloqué jusqu'à leur majorité, avec un taux de rémunération supérieur au livret A et un régime fiscal très incitatif et tout à fait exceptionnel- zéro charge, zéro impôt. Nous attendons 1 milliard d'euros de collecte de ce plan d'épargne avenir climat. Toujours pour mobiliser l'épargne des Français, nous souhaitons aussi que, dans les plans d'épargne retraite et les contrats d'assurance vie, au moins une unité de compte soit obligatoirement consacrée aux investissements verts. Au total, nous voulons mobiliser 5 milliards d'euros d'épargne privée pour le financement de l'industrie verte. Enfin, toujours sur le financement, nous voulons être- je le disais en introduction -le premier pays en Europe à mettre en place un crédit d'impôt pour la production industrielle verte. On en manquait ... Aujourd'hui, quand nous ouvrons des usines comme ACC, ProLogium ou d'autres, nous apportons des subventions- c'est ce qu'a aussi fait l'Allemagne récemment avec Intel. Si nous voulons attirer d'autres investisseurs qui ont besoin de rentabiliser leur investissement sur le long terme et d'avoir de la visibilité, il faut aussi accorder des crédits d'impôt. Je le répète, nous vous proposons, avec ce projet de loi, d'être la première nation en Europe à mettre en place ces crédits d'impôt pour la production industrielle verte. L'intégralité de ce crédit d'impôt, je le précise, sera financée par la réduction de niches fiscales sur les énergies fossiles, conformément à la stratégie que j'ai définie hier de bascule de la fiscalité brune vers la fiscalité verte.

Nous allons donc mettre en place un label d'excellence environnementale européenne, dit triple E, qui doit valoriser les entreprises les plus vertueuses et leur donner un accès privilégié à la commande publique, qui représente 150 milliards d'euros par an. Personne ne peut comprendre que, dans les appels d'offres pour la commande publique, ce soit systématiquement le

Je pense que, à tout point de vue, nous en sortirons gagnants. Je précise également que nous serons la première nation en Europe à réserver le bonus sur les véhicules électriques à ceux qui sont produits dans les conditions environnementales les plus satisfaisantes, c'est-à-dire à des véhicules produits en Europe. Je dois dire qu'il est compliqué, dans un temps de responsabilité budgétaire où l'argent public est rare, de voir que, sur 1,2 milliard d'euros

alors qu'il devrait être attribué sur critère environnemental, en tenant compte des conditions de production. C'est une vraie rupture que nous vous proposons, en réservant ce bonus aux véhicules produits en Europe. Enfin, nous voulons renforcer la formation et la qualification. Nous défendrons plusieurs mesures sur ce sujet comme l'augmentation de 22 % du nombre de places dans les écoles des mines-télécom à l'horizon 2027 et la création de cent écoles de production, toujours à l'horizon 2027.

Nous avons engagé la réindustrialisation : nous vous proposons de l'accélérer et de la verdir. Je suis certain que nous parviendrons à trouver un accord sur ce texte. La parole

je ne veux pas être très long, puisque le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a dit l'essentiel. Je voudrais quand même vous relater quelques événements qui se sont produits non pas ces dernières années, mais ces dernières semaines,

ces résultats du mois qui vient de s'écouler sont avant tout le résultat d'années de travail. Ce sont singulièrement les cinq dernières années qui nous ont permis de retrouver la compétitivité pour le site France.

aujourd'hui à un retour en force de l'apprentissage et à un retour en force des usines. Vous le savez, on ouvre aujourd'hui des usines dans tous vos territoires : dans la Somme, à Nesle ; dans le Doubs, à Allenjoie ; en Saône-et-Loire, à Autun ; en Seine-Maritime, au Havre ; dans la Drôme, à Pierrelatte dans l'Aube, à Sainte-Savine ; dans l'Eure, à Louviers ; dans le Pas-de-Calais, à Auxi-le-Château ; en Ardèche, à Ardoix ; en Gironde, à Saint-Loubès. Partout en France, on rouvre des usines et nous pouvons en être extrêmement fiers.

Notre devoir collectif à toutes et à tous, c'est de construire cette France de 2030 qui donnera à chacun les moyens de faire ce qu'il fait de mieux : inventer, financer, créer, penser, façonner, fabriquer,

veut aussi dire- c'est là l'essentiel de ce projet de loi -que nous avons besoin de foncier, de financements et de simplicité pour l'implantation de projets dans nos territoires. Nous devons poursuivre le changement de mentalité. C'est exactement ce que nous vous proposons dans le cadre de ce projet de loi, qui est le maillon indispensable d'une stratégie de réindustrialisation globale. Au fond, ce texte est un élément essentiel d'un dispositif bien plus large qui prend place dans un environnement de compétition internationale accrue.

un tableau de bord d'automobile en plastique à partir d'une bouteille recyclée, il faut un an de procédure pour que ladite bouteille n'ait plus le statut de déchet. Nous vous proposons de passer dans ce qu'on appelle le « statut implicite

le projet de loi relatif à l'industrie verte, dont nous commençons aujourd'hui l'examen, se donne pour objectif de réindustrialiser la France et de nous donner les moyens de devenir leaders dans les technologies clés de la transition écologique. En accélérant les implantations industrielles, en renforçant la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique, en améliorant le financement de la transition écologique, vous nous promettez, messieurs les ministres, 40 000 créations d'emplois et 23 milliards d'euros d'investissements supplémentaires à l'horizon 2030. Qui pourrait s'opposer à un tel programme ? Soyez-en assurés, messieurs les ministres, nous aurions voulu applaudir des deux mains depuis le temps que nous alertons sur les effets délétères de la désindustrialisation, sur cette sur cette chimère de l'industrie sans usine et de la tertiarisation à tout-va qui a appauvri nos compatriotes, déstructuré nos territoires, atrophié notre recherche et développement et, plus grave encore, qui a mis en péril notre souveraineté et amoindri nos capacités d'adaptation face aux grands défis de demain, au premier chef celui de la transition écologique. Nous sommes d'accord sur les objectifs. Oui, il faut adapter notre industrie à la transition écologique pour nous donner les moyens de tenir nos engagements en matière climatique et de biodiversité. Oui, il faut profiter du puissant catalyseur économique que sont les changements d'usage massifs qui s'annoncent dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'hydrogène et des batteries. Nous aurions donc voulu applaudir votre texte, mais force est de constater qu'après avoir suscité l'enthousiasme il a provoqué la déception. Le texte est consensuel, mais bien en deçà des objectifs affichés ; il contient des mesures techniques qui sont sans commune mesure avec le redressement industriel qu'il nous faut opérer.

vouloir décarboner l'industrie et soutenir les technologies des secteurs du développement durable. Mais, en réalité, au-delà des emblématiques mâts d'éoliennes et des giga-usines de batteries, l'industrie la plus verte n'est-elle pas surtout l'industrie qui produit en France,

Les grands défis de demain, nous les affronterons aussi avec, hélas, notre industrie de défense, ou avec notre industrie pharmaceutique, que vous avez citée, pour vaincre les nouvelles menaces épidémiologiques. Si la crise sanitaire a eu un mérite, c'est bien celui d'avoir mis au grand jour la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement, y compris dans des secteurs stratégiques. Que prévoit votre texte sur ces sujets ? Le plus gênant dans ce texte n'est pas le flou de son objet ou le caractère disparate des mesures proposées ; c'est son incomplétude. Celle-ci se mesure au nombre d'amendements que nous avons dû déclarer faute de lien avec celui-ci, alors même qu'ils auraient pu profondément enrichir la démarche. Je sais que c'est frustrant et je tiens à vous dire, mes chers collègues, que je partage votre déception.

Qu'est-ce qu'une politique industrielle sans mesures financières et fiscales ? Pas grand-chose, sinon une forme de marketing politique ! Parmi les 40 000 créations de postes promises que j'évoquais tout à l'heure, combien sont supposées découler directement de ce texte ? Nul ne le sait. Les mesures que l'on nous propose vont dans le bon sens, mais elles ne vont pas assez loin, comme en témoignent les dispositions dont la commission des affaires économiques Elles visent à améliorer l'attractivité de la France en remédiant à deux faiblesses bien identifiées, que vous avez évoquées : la limitation des disponibilités foncières et la longueur des procédures administratives d'installation. La question du foncier est fondamentale. En France, deux tiers des intercommunalités déclarent avoir déjà refusé des projets d'implantation économique par manque de foncier. Pour réindustrialiser la France, 16 000 à 20 000 hectares seront nécessaires. Environ la moitié pourrait provenir du recyclage de friches, l'autre moitié requerrait une artificialisation nouvelle. C'est un enjeu majeur La commission des affaires économiques a donc complété les dispositions des articles 5 et 6 visant à faciliter la mobilisation du foncier pour des usages industriels elle a prévu l'identification des friches au sein des schémas de cohérence territoriale (Scot), en complément du pilotage existant aux échelons régional et communal. Elle a permis aux communes de récupérer plus facilement des terrains abandonnés pour y réimplanter de l'industrie. Messieurs les ministres, il y a beaucoup à faire pour redonner la main aux communes sur leur foncier. Les fourches caudines de l'article 40 de la Constitution nous contraignent, mais j'aimerais que vous preniez l'initiative sur des thèmes comme le régime des biens sans maître, ou encore celui des biens en état d'abandon manifeste. Afin de permettre un pilotage des implantations industrielles sur le foncier disponible, la commission a aussi limité, sauf exception, les obligations de dépollution après un usage industriel à ce qui est nécessaire pour un nouvel usage industriel. Elle a également permis au tiers demandeur d'intervenir plus tôt, pour anticiper la réhabilitation des friches. En revanche, la commission s'est opposée à la restriction du champ des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui sont soumises à l'obligation de constituer des garanties financières pour financer la remise en état des sites après cessation d'activité : les collectivités se trouvent souvent bien démunies face à ces friches dont les coûts de dépollution peuvent être faramineux. La simplification et la recherche de la compétitivité ne doivent pas se faire au détriment des collectivités locales. Nous attendons un engagement fort de l'État pour accompagner celles-ci, y compris financièrement. Là encore, il manque à ce texte un volet financier pour le rendre crédible

Compte tenu des enjeux en matière d'emploi, de pouvoir d'achat et de souveraineté, prendre le risque de passer à côté de projets industriels par manque de foncier dans les territoires, alors qu'ils représentent si peu d'hectares en valeur absolue, serait une folie. Or deux tiers des EPCI ont refusé des implantations économiques faute de foncier ! Le nouvel article Le nouvel article 9 exclut donc du décompte du ZAN toute artificialisation induite par des implantations industrielles concourant à la transition écologique et à la souveraineté nationale, quelle que soit leur taille. Il s'agit d'une mesure cardinale pour renforcer notre attractivité, car le foncier est la première ressource que recherchent les industriels pour s'implanter, vous l'avez dit monsieur le ministre. Il ne s'agit pas ici d'opposer l'industrie à l'écologie ! Nous parlons ici de faciliter l'implantation d'industries qui contribuent à la transition écologique.

En ce qui concerne le second vecteur d'accélération mobilisé dans ce projet de loi, à savoir l'accélération des procédures administratives, nous avons travaillé dans deux directions : d'une part, permettre à l'ensemble de la chaîne de valeur de bénéficier de ces mesures d'accélération, en élargissant le champ des bénéficiaires de la procédure de déclaration de projet aux activités de recherche et développement et aux sous-traitants d'autre part, mieux associer les collectivités territoriales à la nouvelle procédure accélérée créée à l'article 9. L'acceptation locale est essentielle au succès du déploiement d'implantations industrielles dans les territoires.

mais l'État et les collectivités ont travaillé en parfaite symbiose, ce qui est gage de fluidité et d'accélération. C'est ce que nous devons rechercher, plutôt que de court-circuiter les collectivités locales donnez des moyens aux services déconcentrés de l'État pour mieux accompagner les porteurs de projets dans les territoires, pour mieux outiller les collectivités, pour coconstruire avec elles ces projets stratégiques et en assurer le pilotage, avec toutes les parties prenantes ! C'est ainsi que nous gagnerons, ensemble, la bataille de la réindustrialisation. Cela étant dit, la commission partage l'objectif de permettre l'installation rapide de très grands projets stratégiques. Dans un esprit de responsabilité, elle a donc conservé la nouvelle procédure créée à l'article 9, mais elle l'a profondément réformée, pour redonner l'initiative aux collectivités. Nous avons ainsi dû forcer l'État à dialoguer avec les collectivités, puisque vous ne le prévoyiez pas. Évidemment, nous avons prévu qu'aucune évolution des documents d'urbanisme ne pourrait intervenir sans l'accord des collectivités concernées. Très bien ! C'est une évidence qu'il convenait de rappeler, tout comme la nécessité d'assurer une vraie consultation du public.

Celui-ci, messieurs les ministres, est un patchwork de mesures très techniques et parfois cosmétiques qui devraient, à notre sens, avoir peu d'effet sur les émissions de gaz à effet de serre et ne contribuer qu'à la marge à la réindustrialisation de la France. À l'inverse, certains leviers restés à l'écart de ce texte, et qui semblent plutôt relever du pouvoir réglementaire, pourraient avoir un impact bien plus grand au regard de cet objectif ; je pense par exemple à l'encadrement des délais contentieux en matière d'implantations industrielles. Afin d'améliorer ce texte imparfait, notre commission a donc adopté 34 amendements dans un triple objectif : garantir l'intégrité environnementale du projet de loi, corriger des dispositifs qui n'atteignent pas leur cible, enfin, assurer la sécurité juridique d'un texte imprécis. Je commencerai par le premier volet, à savoir les modifications visant à garantir l'intégrité environnementale du projet de loi. La réindustrialisation ne doit pas se faire au détriment du principe pollueur-payeur. La commission a ainsi rétabli l'obligation de garanties financières pour assurer la réhabilitation des friches industrielles, que le Gouvernement proposait de supprimer à l'article 6. Notre commission a également souhaité préserver le principe et la qualité de la participation du public, gage de l'acceptabilité des projets d'industrie verte. Nous avons ainsi aménagé, par plusieurs amendements, la modernisation de la procédure de consultation proposée par le Gouvernement aux articles 2 et 3, pour assurer un meilleur équilibre entre démocratie environnementale et réindustrialisation. La compensation des atteintes à la biodiversité, prévue à l'article 7, a été modernisée et sécurisée : notre commission a souhaité mieux distinguer les notions de « restauration » et de « renaturation », d'une part, de « compensation », d'autre part.

modifications visant à corriger des dispositifs qui n'atteignent pas leur cible. À l'article 13, afin de garantir que les organisations assujetties respecteront leur obligation d'établir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (Beges), notre commission a relevé les sanctions administratives applicables et a supprimé l'exclusion facultative des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession en cas d'irrespect, proposée par le Gouvernement. Par cohérence, la possibilité de mobiliser des critères qualitatifs, notamment environnementaux, pour attribuer les marchés publics a été étendue aux contrats de concession. Enfin, notre commission a conforté la consécration juridique de la sortie implicite du statut de déchet, prévue à l'article 4, en proposant une rédaction plus robuste. Le troisième volet comprend les modifications tendant à renforcer la sécurité juridique d'un texte parfois imprécis.

Au préalable, je voudrais exprimer notre regret quant à l'absence de définition de cette notion : l'industrie verte, est-ce seulement les pompes à chaleur, les panneaux solaires, les pales d'éoliennes, l'hydrogène vert ou encore les batteries électriques

En effet, le titre III traduit plutôt deux autres objectifs, sans lien direct avec les enjeux environnementaux : attirer l'épargne privée vers les entreprises non cotées et maintenir la compétitivité de la place de Paris.

L'article 16, quant à lui, crée ce fameux nouveau produit d'épargne réservé aux mineurs, le plan d'épargne avenir climat, dont les fonds devront être alloués au financement de l'économie productive et de la transition écologique. La commission des finances a largement précisé le fonctionnement de ce produit,

entreprises, ce qui soulève un certain nombre de difficultés. Ainsi, le financement d'activités non cotées par des dispositifs qui peuvent être fermés à tout moment après une certaine durée de détention soulève des problèmes de liquidité. Recourir à la seule valeur estimative n'est pas protecteur

pour pallier l'absence d'argent public pour le financement de la transition écologique et le soutien au tissu industriel, elle est en revanche très circonspecte sur l'efficacité des dispositifs proposés. Le Gouvernement escompte 5 milliards d'euros de collecte, ce qui est très loin des enjeux financiers de la transition environnementale. En 2021, les investissements climatiques ont représenté en France, toutes origines confondues, 84 milliards d'euros. Décarboner les quatre secteurs de l'industrie lourde à l'origine de près de 10 % des émissions nationales de gaz à effet de serre nécessite de mobiliser 14 milliards d'euros chaque

Quel contraste, cependant, avec le présent projet de loi ! Alors que celui-ci nous est décrit comme un moyen de « privilégier une commande publique responsable », force est de constater que, si les mesures proposées ne sont pas inutiles,

de rappeler aux acheteurs publics qu'ils ont la faculté de prendre en compte des critères environnementaux lors de l'appréciation de l'offre économiquement la plus avantageuse. S'agissant de l'article 12,

il est régulièrement proposé au législateur d'insérer dans le code de la commande publique de nouveaux motifs d'exclusion de la commande publique. Ce fut par exemple le cas lors de l'examen de la loi Climat et résilience. approche, qui peut se comprendre, est d'inciter les entreprises à respecter des obligations de nature économique, sociale, éthique, ou encore environnementale, en utilisant la commande publique comme outil incitatif. cette multiplication des motifs d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession soulève un enjeu d'effectivité et d'application du droit au regard de leur très faible utilisation par les acheteurs publics. (Ugap), la principale centrale d'achats publics, m'a indiqué, lors de son audition, que l'on ne mettait jamais en oeuvre ces dispositifs d'exclusion des contrats publics, qui ont pourtant fleuri dans le code de la commande publique en l'espace de quelques années. C'est pourquoi, lors de votre audition par les quatre rapporteurs, monsieur le ministre Le Maire, je vous ai interrogé sur les instructions que vous envisagiez de donner afin de rendre enfin applicables ces pans entiers du droit de la commande publique, en sensibilisant davantage les acheteurs publics sur les facultés d'exclusion que leur offre le code de la commande Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour donner suite à l'engagement que vous avez alors pris devant nous de mettre en oeuvre des actions de communication afin d'inciter les acheteurs publics à avoir davantage recours aux motifs d'exclusion des contrats publics que le Gouvernement soumet fréquemment à nos votes. Nonobstant ces réserves et du fait de notre choix délibéré de faire confiance à cet engagement du Gouvernement, la commission des lois a adopté une position constructive sur l'article 12. Sans pour autant nous illusionner sur la portée réelle de cet article, nous l'avons en effet approuvé, en considérant qu'il participera à renforcer l'effet de signal qu'il a pour les entreprises. conformément à la position constante du Sénat, consistant à limiter le recours aux ordonnances aux cas les plus justifiés, la commission des lois a adopté deux amendements à cet article, visant à mieux encadrer le périmètre de l'habilitation à légiférer par ordonnance demandée par le Gouvernement

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis 2020, nos défaillances en matière industrielle, qui ne datent pas d'hier, sautent aux yeux.

Nous verrons ce qui ressort de nos prochains échanges. Je sais que chacun tient à ce que la transformation écologique de la France soit une réussite. Réindustrialiser notre pays constitue le meilleur vecteur pour décarboner des pans entiers de nos productions, grâce à la mise en oeuvre de technologies bénéfiques au développement durable.

Le projet de loi ouvre un autre chemin pour financer cette transition : la mobilisation des capitaux privés. Dès février 2021, j'ai proposé un dispositif de mobilisation de cette épargne pour financer les projets industriels dans nos territoires. Épargne privée, assurance vie, plan d'épargne retraite, capital-risque, capital investissement, etc. : les leviers sont nombreux qui peuvent contribuer à l'effort de financement. Cette approche non coercitive présente deux avantages elle permet de ne pas imposer davantage les Français ; d'autre part, elle stimule l'innovation dans la transition en contribuant à « dérisquer » les investissements les plus essentiels.

Tandis que certains n'ont eu de cesse de pousser à une mondialisation ultralibérale de l'économie, les écologistes appellent, depuis de nombreuses années, à rétablir notre souveraineté industrielle et à engager une relocalisation de notre industrie, en particulier pour les productions stratégiques essentielles pour l'environnement, la

de vouloir réindustrialiser sans prendre en compte l'ensemble de ces impacts. Ce texte, dans son ensemble, n'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Il ne contient pas de réelles mesures permettant de parvenir à une réindustrialisation décarbonée et résiliente, qui s'inscrirait dans une logique de sobriété et qui occasionnerait la création d'emplois verts dans les territoires. La décarbonation, qui est tant mise en avant, est de plus quasi absente du texte. Les voies et les moyens pour l'atteindre ne sont pas définis ou sont renvoyés au domaine réglementaire.

Réindustrialiser, c'est d'abord préserver, adapter et régénérer ces tissus industriels territoriaux. Je pense par exemple à Photowatt, entreprise victime du chinois

ne lésine pas sur les mesures régressives concernant les règles environnementales et sur l'affaiblissement du processus de consultation démocratique, sous couvert bien sûr d'accélération des procédures

Nous saluons tout de même une avancée intervenue en commission, grâce à l'adoption de notre amendement visant à créer des projets territoriaux d'industrie circulaire, à l'image des projets alimentaires territoriaux (PAT). La commande publique doit, quant à elle, être plus exemplaire en matière de responsabilité environnementale. Nous ferons des propositions pour renforcer l'ambition du texte en ce sens. Fort heureusement, le drame de la réindustrialisation à marche forcée contre les collectivités est évité. La tentative de recentralisation, contraire au principe de libre administration des collectivités, a avorté,

années de désindustrialisation et d'appauvrissement de régions entières, dont la richesse et l'organisation de la vie en société s'articulaient autour de l'industrie- cet idéal de production qui alimente le progrès technique et le développement de toute l'économie nationale.

menant une politique de l'offre ambitieuse, qui a indubitablement attiré les investisseurs puisque, depuis quatre ans, la France est le pays européen qui reçoit le plus d'investissements

Elle doit tenir compte des enjeux propres à notre époque : la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation à ses conséquences. C'est pourquoi le texte que nous allons examiner est une composante fondamentale d'une politique industrielle ambitieuse, orientée vers l'objectif de décarbonation et visant à faire de la France un pays leader

le cas du crédit d'impôt pour les investissements dans les industries vertes. À cela s'ajouteront des mesures réglementaires, telles que l'introduction d'un label d'excellence environnementale pour soutenir les entreprises les plus vertueuses, ou encore le conditionnement du bonus écologique à l'empreinte environnementale des véhicules électriques. Par ailleurs, des investissements substantiels ont été déployés depuis 2017, dans le cadre notamment des plans France Relance et France 2030. Des sommes considérables ont ainsi été mobilisées pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés-

en oeuvre de procédures plus efficaces, dans des conditions attractives, ce projet de loi nous permettra d'accélérer les décisions d'investissement et de renforcer notre base industrielle.

je vous remercie

dispositifs financiers, comme le suggère Jean Pisani-Ferry, et instaurer une fiscalité climatique spécifique. Dans ce contexte, je reprends à mon compte les propos du professeur Pierre Veltz, qui appelle, « dans une perspective positive, à construire le récit d'une économie désirable ».

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, décarboner notre industrie et créer les conditions de notre souveraineté technologique constituent des objectifs dont la réalisation revêt un caractère d'urgence. Le réchauffement climatique ne cesse de nous le rappeler au gré des phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient et qui, depuis quelques années, sont devenus la norme. L'enjeu est colossal. La question industrielle est au croisement de tous les défis- sociaux, environnementaux, technologiques -et les crises mondiales qui se succèdent nous l'ont démontré.

Le levier utilisé par les États-Unis n'est donc ni la liberté d'entreprendre ni même celle d'investir. C'est bien le soutien à la consommation des ménages qui est au coeur de ce plan, ainsi que l'octroi d'aides publiques sous réserve de l'achat de produits issus du territoire. À court terme, les États-Unis débloquent des aides d'État ; à long terme, ils s'assurent une souveraineté technologique, industrielle, et énergétique. La réponse européenne a été timide. Si la

Comment ce texte permettra-t-il de conserver la production en France, d'empêcher les délocalisations et la diminution des activités dites « moins rentables », comme la recherche et le développement ?

Or, sans formation, notre pays ne développera aucun des savoir-faire techniques et technologiques qui conditionnent toute reprise industrielle. Quant aux travailleurs et aux travailleuses, que ce gouvernement a malmenés en leur imposant une réforme

contrôle à lui seul les trois quarts de la production mondiale de batteries aux ions de lithium utilisées dans les voitures électriques. Ces faits sont alarmants. Le poids de l'industrie dans l'économie française a été divisé par deux depuis 1970. Il se stabilise depuis six ans autour de 12 % du PIB, alors que ce taux atteint 23 % en Allemagne. Durant les cinq dernières années, l'industrie française a créé 90 000 emplois salariés et l'on dénombre 80 créations nettes d'usines en France en 2022. Ces prémices d'un renouveau industriel doivent être encouragées et être conciliées avec de véritables stratégies de développement durable. Le projet de loi que nous examinons est d'abord un texte technique, qui vise à renouveler le cadre juridique de manière opportune.

Au Sénat, le 31 mai dernier, vous affirmiez, monsieur le ministre Le Maire, que ce projet de loi était « décisif pour accélérer la réindustrialisation de notre pays et réussir la transition écologique Pourtant, au vu des travaux du Sénat, si ce projet de loi va dans le bon, ses contours sont flous et il manque d'une vision globale de la réindustrialisation. En effet, il se restreint aux industries du, qui ont été citées. Se focaliser sur ces technologies, qui sont certes importantes, c'est faire l'impasse sur les nombreuses autres industries stratégiques qui contribuent elles aussi à la décarbonation de notre économie et aux défis de production. Je pense aux filières de recyclage et de réemploi et aux matières premières biosourcées, qui sont incontournables dans un monde où les ressources en matières premières sont finies.

contradictions qui sont préjudiciables aux actions et à la bonne compréhension locale de ces dispositions sur le terrain. En matière d'industrie, une vision globale, ambitieuse et consolidée s'impose sur l'ensemble des secteurs, mais aussi dans la durée. rien n'est dit sur l'innovation et la recherche ; rien n'est dit sur la formation et le défi du recrutement ; rien non plus concernant l'avenir de nos PME et entreprises

également indiqué ceci : « Chaque relocalisation contribue à réduire l'impact de nos activités à l'échelle mondiale. L'atteinte de nos objectifs économiques et climatiques passe par une nouvelle étape d'accélération des implantations

souhaitez réduire nos impacts à l'échelle mondiale. Le constat est partagé : la désindustrialisation a eu pour conséquences économiques et sociales, en France, la perte de millions d'emplois, mais aussi d'un savoir-faire et d'une expertise. Pour autant, nous ne pouvons pas reconquérir les marchés n'importe comment. L'état des lieux du réchauffement climatique et les rapports consternants du Giec sur la disparition de milliers d'espèces animales et végétales nous obligent à faire preuve de raison et d'anticipation. Nous avons la responsabilité de faire face à ces défis.

ailleurs, comment connaître l'impact carbone lorsque les évaluations et les labels ne sont pas identiques ? À l'heure où les groupes ont compris l'intérêt d'une image verte, comment lutter contre le ? Il est primordial de faire évoluer les marchés publics et de les affiner.

Côté fiscal, la France enregistre un déficit commercial sur les biens de 160 milliards d'euros et accumule chaque année près de 150 milliards d'euros de taxes, impôts et cotisations supplémentaires par rapport à ses voisins de la zone euro- sans parler des normes. Difficile, dans ces conditions,

avons proposé de créer une procédure continue de consultation du public qui couvre toutes les phases du projet d'infrastructure, sous l'égide d'un garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP). Cette recommandation est adaptable aux projets d'implantation d'industrie verte, car les réunions publiques que vous citez ne relèvent en rien de la coconstruction. En général, les projets sont déjà ficelés lorsqu'ils sont présentés aux habitants, lesquels le savent bien. Messieurs les ministres, vous l'avez compris, de nombreuses questions demeurent à la lecture de ce texte. J'espère que le débat que nous allons avoir nous aidera à y voir plus clair. La parole

j'ai été frappé par l'une de ses remarques, qui illustre à mon sens les limites du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Il pointait le paradoxe de ce texte. d'un côté, le Gouvernement dit vouloir accélérer les implantations industrielles et affirme, à cet égard, se préoccuper de la mobilisation du foncier industriel. D'un autre côté, loi ne comporte pas un mot sur l'objectif ZAN, qui, de l'avis d'une large majorité des acteurs locaux, constitue pourtant le principal obstacle à la disponibilité du foncier en France. Cette anomalie me laisse perplexe, d'autant plus qu'elle ne fait pas figure d'exception dans ce texte selon moi inachevé. Une fois de plus, l'exécutif raisonne par petits bouts, sans chercher de cohérence globale.

pourquoi réserver ces objectifs majeurs à un seul type d'activité ? Pourquoi réserver la simplification des normes et des procédures à certaines entreprises ? Je pense à l'immense majorité des entreprises dans nos territoires : les PME, et ses petits patrons, qui n'ont ni les moyens de gérer la complexité ni la chance de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Faute d'une vision systémique de la simplification administrative, pourtant prônée par les auteurs de ce projet de loi, nous manquons, une fois de plus, notre cible. Il ne faut pas seulement simplifier la construction des usines, mais englober toute la chaîne de valeur dans une démarche de simplification. Sinon, les PME sous-traitantes des que les ministres ne manqueront pas d'inaugurer seront toujours engluées dans la complexité de la délégation aux entreprises du Sénat, j'ai présenté la semaine dernière un rapport d'information sur la simplification des normes et des règles applicables aux entreprises. Mes collègues rapporteurs Gilbert-Luc Devinaz et Jean-Pierre Moga et moi-même martelons sans relâche cet effrayant diagnostic le fardeau normatif coûte 60 milliards d'euros par an, soit 3 % de notre PIB, dont 28 milliards d'euros rien que pour nos ETI. Nous devons réagir vite et collectivement. Dans le respect des prescriptions environnementales et des équilibres sociaux, notre effort de simplification doit impérativement être pensé de façon systémique, constante, déterminée et, surtout, pour toutes nos entreprises périmètre de ce texte, qui regorge de mesures très techniques et très ciblées est, au contraire, beaucoup trop restreint. C'est pourquoi les amendements que je défendrai visent à étendre le processus accéléré d'implantation à toutes les PME qui participent, de façon directe ou indirecte, aux chaînes de valeur des secteurs concernés par le projet de loi. Messieurs les ministres, je compte sur votre bon sens pour émettre sur eux un avis favorable. Seule une acception large permettra de transformer l'ensemble de nos chaînes de production. Seule une démarche systémique aura un véritable impact sur la décarbonation de notre économie. La parole

ce changement confronte notre espèce, et la nature, à leurs dernières extrémités ; parce qu'il nous approche du bord de nos modes de vie, de nos ressources ; parce qu'il nous pousse tout au bout des contradictions de nos économies centrées sur la consommation », écrivait la semaine dernière

pluriannuelle de l'industrie, voire de l'écologie, à revoir tous les cinq ans, pour nous adapter efficacement à ce qui vient. De plus, quel sera le coût réel de notre production en matière de dégradation de la santé et d'effondrement de la biodiversité ? une industrie verte doit être l'occasion de prévoir la satisfaction de nos besoins essentiels et de remettre à l'honneur- pourquoi pas -la manufacture et l'artisanat, qui sont les seules véritables expressions de l'industrie, au sens de l'inventivité humaine. Autrement, l'industrie verte ne sera qu'un avatar sémantique de plus.

et deviennent instantanément, en arrivant en Afrique, des déchets. Nous avons une énorme responsabilité. Comment expliquer que le chapitre dédié à l'économie circulaire soit si pauvre ? C'est dommage

texte en commission a permis d'obtenir des avancées. À l'article 2, nous avons ajouté à la consultation numérique la consultation par voie postale, qui est absolument indispensable, sachant qu'un Français sur trois est concerné par l'illectronisme.

Vous l'aurez compris, messieurs les ministres, nous attendons davantage, bien davantage, car les défis sont colossaux. Réindustrialisons, mais faisons-le bien : l'argent public doit être mieux utilisé, et, surtout,

devait être amorcée par le projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Mais cette révolution aura-t-elle bien lieu ? Attendu comme la pierre angulaire d'une nouvelle dynamique industrielle, ce projet de loi répond à des objectifs louables, que tous, sur ces travées, nous partageons. La réindustrialisation de notre pays et la décarbonation de notre industrie doivent permettre à la France de devenir un champion international des technologies décarbonées, tout en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle planétaire, la concurrence fait rage ; nous devons être à la hauteur du défi. Le protectionnisme économique chinois et les milliards de l'sont autant de symboles de ce contexte international concurrentiel, d'une densité inédite. Les enjeux sont clairement identifiés et les besoins connus. Nous ne pouvons que saluer les mesures de simplification salutaires qui sont introduites par ce texte. Elles feront chuter le délai réel d'implantation des usines sur notre territoire. En effet, cependant que l'Allemagne met entre quatre et douze mois pour implanter une usine, ce projet de loi doit nous permettre de réduire ce délai de

Pourtant, un fossé regrettable existe entre l'ambition affichée par le Gouvernement et le contenu de ce texte. Nous restons au milieu du gué quant à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de nos industries. Texte technique, ce projet de loi relatif a tout du fourre-tout et ne constitue en rien la révolution attendue. Aux côtés de nos rapporteurs Laurent Somon, Fabien Genet, Jean-Yves Roux et Christine Lavarde, que je remercie profondément de leur engagement, nous avons oeuvré pour enrichir ce texte, le sécuriser et en faire un véritable atout pour notre industrie, plutôt qu'un simple signal pour les investisseurs étrangers. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et le Sénat ont pris toute leur part pour ajuster ce texte. La protection du principe pollueur-payeur, la préservation du rôle primordial de la participation du public au sein de la procédure d'autorisation environnementale ou la création de projets territoriaux d'industrie circulaire sont autant de garanties apportées par le Sénat en matière environnementale.

aux plus petites collectivités permettra aux élus de s'appuyer sur un outil juridique innovant afin de verdir, à leur échelle, la commande publique. En effet, le verdissement de la commande publique ne doit pas être l'apanage des grosses collectivités. Il s'agit d'un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs publics. Texte nécessaire, ce projet de loi ne répond donc que partiellement aux attentes majeures qu'il avait suscitées. Pourtant, en responsabilité, le Sénat l'a enrichi et ajusté de manière significative afin de permettre

le foncier est la première aménité que recherchent les industriels. Si nous ne le leur fournissons pas, toutes les autres mesures que nous prendrons pour encourager les implantations d'usine en France seront vaines. Je rappelle que, selon une enquête menée l'an dernier, deux tiers des intercommunalités ont refusé des projets d'implantation économique ou subi des déménagements d'entreprise par manque de foncier économique.

elle devrait inclure l'ensemble des projets industriels qui favorisent la transition écologique. Monsieur le ministre Le Maire, vous avez exprimé, lors de votre audition au Sénat le 31 mai dernier, votre souhait, à titre personnel, d'exempter les grands projets industriels de l'objectif du ZAN, en affirmant laisser « à la sagesse des parlementaires le soin de savoir si on exempte du ZAN uniquement les projets portant sur l'industrie verte répondant à la définition des actes européens [ ...] ou si nous élargissons à d'autres projets industriels dont nous estimons qu'ils favorisent aussi la transition écologique Dans sa sagesse, la commission des affaires économiques et son rapporteur Laurent Somon- dont je salue le travail -ont tranché : le nouvel article 9 exclut l'ensemble des installations industrielles « concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale » du décompte du ZAN- qu'il s'agisse du décompte à l'échelon local, régional

une autre vision semble s'exprimer à l'Assemblée nationale, où la commission des affaires économiques a adopté la semaine dernière un amendement à notre proposition de loi visant à mutualiser entre régions l'artificialisation des grands projets industriels, au lieu de l'exclure totalement du décompte. Pis encore, le texte le texte issu de la commission prévoit que ce seront non pas tous les projets industriels d'intérêt national qui seront exclus du décompte régional du ZAN, mais seulement ceux d'entre eux qui seront désignés par décret-

texte voté par le Sénat, qui prévoyait que les collectivités locales, sous la houlette des régions, puissent se prononcer sur les grands projets industriels. C'est le seul moyen pour que celles-ci aient leur mot à dire sur les projets qui profiteront de l'exemption de ZAN, qui les concerne tout de même au premier chef ! La commission n'a donc fait que donner aux collectivités les garanties que le ministre Béchu s'était engagé,

mais la maîtrise des technologies vertes- le tout par les territoires.

D'autre part, les auditions ont démontré que les acheteurs publics avaient déjà beaucoup de difficulté à s'approprier la faculté que leur ouvre le code de la commande publique d'exclure des candidats. Les contrôles sont succincts et la plupart des acheteurs publics n'ont pas les ressources suffisantes pour procéder à des vérifications en profondeur. Le contrôle des fournisseurs risquerait donc, au mieux, de ne pas être fait, au pire, de constituer une charge administrative très lourde pour les acheteurs publics. Quel est l'avis

ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. Cette disposition, qui pourrait constituer un puissant levier au service de la réindustrialisation la réindustrialisation verte et de la souveraineté économique de l'Europe, est très peu utilisée par les acheteurs, à qui n'ont jamais été clairement précisés les cas dans lesquels ils pourraient concrètement y recourir. Seul cas connu, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) en a recommandé l'usage pour l'achat d'équipements de protection individuels en décembre 2021. Cet amendement vise donc à ce que les services de l'État puissent préciser aux acheteurs les conditions d'application de cet article, et notamment indiquer si ces dispositions peuvent s'appliquer à d'autres secteurs, par exemple en matière de production d'énergie renouvelable comme les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. La

il faut clarifier les choses sur la commande publique pour que la souveraineté économique européenne soit indirectement bénéfique pour la souveraineté économique de la France.

En effet, pour un certain nombre de marchés, par exemple les lignes à haute tension, du fait de la rareté de l'offre, il est plus pratique pour RTE d'émettre un seul lot plutôt que de faire de l'allotissement.

l'amendement n° 329 rectifié permettrait aux autorités adjudicatrices de procéder à des appels d'offres lors desquels la présentation de variantes serait autorisée, ce qui va totalement à l'encontre de l'article L. 2151-1 du code de la commande publique.

aux marchés de réseau ont une raison d'être que le Sénat a toujours défendue, à savoir garantir l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. Les dérogations que souhaite instaurer le Gouvernement auront mécaniquement pour conséquence de favoriser les plus grandes entreprises, qui sont mieux à même

Qui plus est, le chevauchement de deux dispositifs qui ne sont pas liés instaure une ambiguïté quant aux finalités et à l'application de cet article du code de la commande publique. En outre, la rédaction de cet amendement semble beaucoup trop large, puisque la notion de « procédé industriel » n'est définie nulle part dans le code de la commande publique. Notre collègue souhaite notamment viser les marchés de « fournitures [ ...] qui intègrent des procédés industriels

de l'aménagement du territoire ? Cet amendement me semble satisfait. Le Spaser, qui définit la stratégie d'achat durable des plus grands acheteurs publics, peut d'ores et déjà faire la promotion de l'économie de la fonctionnalité.

n° 52 rectifié. Portés par les technologies du numérique, mais aussi par des usages multimodaux, les services de la mobilité agissent au service de la transformation des pratiques de mobilité et de la promotion de nouveaux comportements vertueux. Alors que le champ d'application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables est élargi et clarifié, cet amendement vise à intégrer aux objectifs de politique d'achat des prérogatives en termes de transition des mobilités.

de mobilités bas-carbone et de repenser nos modèles économiques. Les mobilités actives et partagées constituent un vecteur de la décarbonation des transports. Nous disposons là d'un levier majeur pour répondre aux défis de la transition écologique et d'une plus grande accessibilité aux solutions de mobilité durable. Afin d'accompagner les acteurs publics dans cette démarche, les mobilités partagées, douces et actives peuvent agir en faveur de la transformation des pratiques de mobilité et de la promotion de nouveaux comportements plus vertueux. cet amendement vise à compléter les dispositions relatives au schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables dans le but d'inscrire la politique d'achat dans une démarche de transition vers les mobilités partagées et actives. Quel est l'avis de

Je rappelle qu'il s'agit de mesures de vigilance propres à identifier les risques d'atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, comme les activités des sous-traitants

du territoire ? L'exclusion facultative des candidats n'ayant pas respecté leur obligation d'établir un plan de vigilance a été introduite par la loi Climat et résilience de 2021, sur l'initiative de la commission Sénat. Transformer ce motif d'exclusion facultatif en motif d'exclusion obligatoire ne me semble pas pertinent. Je rappelle que les motifs d'exclusion de plein droit s'appliquent pour des infractions particulièrement graves, par exemple au titre du code pénal- participation à une organisation criminelle, corruption, infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes

du territoire a supprimé cette possibilité au profit du renforcement des sanctions en cas d'absence d'établissement du Beges. À nos yeux, l'un n'empêche pas l'autre. Aussi proposons-nous de rétablir cette exclusion qui, rappelons-le, est une obligation légale pour les 5 000 acteurs privés et publics concernés. Le Beges permet d'élaborer un diagnostic précis des émissions de gaz à effet de serre. Il prend en compte les émissions directes liées à l'activité de l'entreprise et les émissions indirectes liées à la production d'énergie. Il permet aux entreprises et établissements concernés d'identifier les grands postes d'émission et les leviers de réduction de leurs émissions de CO2 dans le cadre d'un plan de transition. Dans la perspective de l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050, il est essentiel que les entreprises s'emparent enfin de cet outil. En effet, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, seuls 53 % des entreprises respectent leurs obligations sur ce point- et encore s'agit-il des chiffres les plus optimistes. Pour une meilleure efficacité et pour respecter l'égalité de traitement entre les candidats, nous demandons le rétablissement de la mesure prévue dans le projet de loi initial en proposant que cette règle soit obligatoire et non une simple faculté, tout en maintenant le renforcement des sanctions pour les entreprises contrevenantes proposé par la commission

pas cette obligation. Par conséquent, utiliser le levier de la commande publique pour la faire appliquer serait une bonne idée.

rempli ses obligations au titre du bilan d'émissions de gaz à effet de serre. C'est à la fois très respectueux des libertés des collectivités locales et très responsabilisant.

dix ans après son entrée en vigueur, 65 % des presque 5 000 organisations assujetties n'ont pas respecté leur obligation de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre.

menées par la commission de l'aménagement du territoire, il est apparu que ces leviers d'exclusion des procédures de passation des marchés publics et de contrats de concession, qu'ils soient de plein droit ou facultatifs, étaient très peu efficaces. Concrètement, les acheteurs publics se contentent souvent d'une déclaration sur l'honneur pour effectuer les vérifications et appliquer les motifs d'exclusion des procédures de la commande publique.

Parmi les différents outils dont dispose la commande publique, les variantes environnementales, solutions alternatives et vertueuses à l'initiative des entreprises, constituent aujourd'hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs. cet amendement vise à faciliter la présentation de variantes environnementales au sein des marchés publics, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire écologique. Ces dispositions entreront en vigueur à partir de la date à laquelle les acheteurs seront tenus d'intégrer un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales des offres, conformément à l'article 35 de la loi Climat et résilience. Ce changement de paradigme dans l'utilisation des variantes s'inscrit parfaitement en cohérence avec l'Agenda 2030, qui fait de la promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics un enjeu majeur, tout comme avec le plan national pour des achats durables 2022-2025. L'amendement

En favorisant un investissement écologique et responsable, les collectivités font le choix d'une commande publique vertueuse. La diffusion de ces bonnes pratiques doit servir de fer de lance pour lancer un nouveau dogme, celui d'un verdissement progressif de la commande publique.

au service au mieux d'une action isolée, au pire du. Alors que nous n'avons jamais été aussi proches d'un point de non-retour, les acheteurs publics peuvent encore se passer de la prise en compte des conséquences climatiques et environnementales de leur commande ! L'offre économiquement la plus avantageuse sert à discriminer les autres offres au profit de la meilleure. Elle est aujourd'hui définie par la voie réglementaire. Ce projet de loi souhaite accélérer la prise en compte des critères environnementaux dans le choix des offres déjà planifiées pour 2026 par la loi Climat et résilience. Aussi, je propose d'inclure systématiquement au moins un critère environnemental ou social. La meilleure offre est celle dont le coût pour la planète est le plus faible. C'est devenu une évidence, mes chers collègues. Ne passons pas à côté de cette ambition pour nos industries vertueuses et pour notre planète.

adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s'agir, par exemple, de la qualité de l'offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes. La proposition de règlement pour une industrie « zéro net » établie par la Commission européenne prévoit que les pouvoirs adjudicateurs et les entités compétentes d'un marché public, la contribution des offres à la durabilité et à la résilience en fonction d'une série de critères. En France, selon l'article R. 2152-7 du code de la commande publique, modifié par le décret du 2 mai 2022,

de se tourner vers l'option écologique la mieux-disante, dès lors que les caractéristiques techniques des différentes offres présentent des performances finales équivalentes. L'objectif est bien d'inciter davantage de collectivités territoriales à s'interroger sur leur stratégie d'achat et à mieux intégrer les enjeux environnementaux.

soumissionnaire. Le Gouvernement propose que les critères environnementaux et sociaux puissent figurer en sus du critère économique. Ce serait une possibilité, mais en aucun cas une obligation.

rectifié et 227 ont pour objet d'anticiper son entrée en vigueur tout en imposant la prise en compte de plusieurs critères qualitatifs dans l'attribution du marché ou du contrat de concession.

ces sept amendements. Le droit européen et le code de la commande publique prévoient que les marchés publics soient attribués selon des critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

que d'adopter ici un texte qui serait contraire au droit en

Je ne crois pas que la prise en considération par l'acheteur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

en compte des critères environnementaux pour l'attribution d'un contrat de concession, qui engloberaient l'ensemble de la chaîne de production et le cycle de vie du produit. Les critères environnementaux permettant d'attribuer un contrat de concession sont librement arrêtés par les acheteurs publics. Nul besoin de préciser que les critères pris en considération par l'acheteur englobent l'ensemble de la chaîne de production et le cycle de vie du produit. De surcroît, ces critères environnementaux, qui pourront être intégrés, devront avoir un lien avec l'objet du contrat de concession, comme l'exige le droit européen. Il n'est donc pas certain que des critères environnementaux englobant l'ensemble de la chaîne de production et le cycle de vie du produit répondent systématiquement à cette condition. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable

En effet, de telles décisions ne prennent pas en compte les externalités environnementales liées au transport sur des milliers de kilomètres, ce qui est difficilement conciliable avec les engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et les efforts à entreprendre pour y parvenir.

Dans le prolongement de mon précédent amendement pour une commande publique toujours plus ambitieuse, cet amendement vise à protéger notre industrie nationale et européenne de produits et matériaux de construction. Le développement des circuits courts est crucial dans la réduction des émissions liées aux transports, participe de la valorisation de nos entreprises et de nos industries

en intégrant de nouveaux critères dans la commande publique. La production d'énergies renouvelables repose sur des processus industriels de fabrication technique et des équipements à fort impact carbone et environnemental. Les entreprises françaises et européennes qui produisent sur notre sol ces composants nécessaires à la création des dispositifs de production d'énergie doivent être les premières bénéficiaires de la commande publique. Afin de garantir une souveraineté énergétique française et européenne durable et propre, il est urgent de donner la priorité aux solutions françaises et européennes à l'importation. C'est pourquoi cet amendement tend à intégrer de nouveaux critères dans la commande publique afin de favoriser les filières françaises de l'industrie verte en cohérence avec l'article L. 2514-2 du code de la commande publique. achats. Monsieur le rapporteur pour avis, et un critère portant sur la qualité de l'offre et un critère relatif au prix ou au coût. Il n'est pas possible de prévoir la seule prise en compte des critères environnementaux ou sociaux, y compris pour des marchés ayant trait à l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable

Concrètement, il s'agit d'adapter les obligations instaurées par la loi d'orientation des mobilités de 2019 en matière de renouvellement des flottes de véhicules d'entreprise. Les avantages écologiques, économiques et techniques du rétrofit ne sont plus à prouver. Il contribue notamment à l'amélioration de la qualité de l'air et permet d'anticiper la fin de vie du parc de véhicules thermiques en 2035. Par ailleurs, les véhicules utilitaires légers et les poids lourds utilisés dans l'industrie et dans le secteur du bâtiment roulent encore massivement au diesel et seront donc les plus concernés par la mise en place des zones à faibles émissions Dans ce contexte, le rétrofit constitue une vraie solution, facilement disponible, car cette technologie est pleinement maîtrisée par les constructeurs européens. Enfin, les appels d'offres des marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont conçus pour l'acquisition de véhicules neufs. Or il est indispensable que nos territoires puissent prendre en compte le rétrofit

abaisse le coût d'entrée vers une mobilité plus durable et permet de proposer des véhicules durables, enjeu crucial dans le cadre de la mise en place des zones à faibles émissions. Les appels d'offres des marchés publics ayant pour objet le remplacement de véhicules lourds sont pensés et structurés structurés pour l'acquisition de véhicules neufs. Il est donc indispensable que nous adaptions les modalités d'application de la loi d'orientation des mobilités concernant le renouvellement des flottes d'entreprise dans l'objectif d'accélérer le verdissement du parc automobile, en intégrant cette technologie.

Faut-il en plus de ces dispositions prévoir un objectif spécifique d'acquisition de véhicules « rétrofités » pour les acheteurs publics ?

qui proposent un critère cumulatif aux critères existants de renouvellement des flottes avec des véhicules à faibles ou très faibles émissions et qui ouvrent plus largement le champ des technologies du rétrofit.

qui prévoit que l'État met à la disposition des acheteurs de la commande publique des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût global du cycle de vie des biens. Pour cela, l'État doit doter l'ensemble des parties prenantes des informations nécessaires à la connaissance d'un produit dans son cycle de vie, de sa production à son recyclage. Le coût total d'un produit doit être rendu transparent pour tous les acteurs afin de promouvoir une véritable industrie verte.

Marie-Claude Varaillas. Nous considérons que toutes les aides publiques doivent être conditionnées au respect des critères sociaux et environnementaux. C'est une priorité à l'heure où presque 200 milliards d'euros d'aides publiques sont versés aux entreprises sans aucune contrepartie. l'argent magique n'existe pas : il faut réformer notre système de protection sociale, raboter les retraites, les soins, l'éducation, la formation. En revanche, lorsqu'il est question de défendre l'attractivité

Cet amendement de repli vise à élargir l'obligation d'établir un Beges intégrant le scope 3 aux entreprises de 250 salariés et plus, ainsi qu'à généraliser l'obligation d'un bilan simplifié aux entreprises de 50 salariés au moins. Actuellement, le bilan carbone requis se limite aux émissions de scope 1, c'est-à-dire aux émissions directes liées à la production du produit, sans exigence de réduction alignée alignée sur les objectifs de l'accord de Paris. C'est insuffisant. Comme le souligne l'Ademe, la décarbonation de nos activités à tous les niveaux de la société est devenue un mot d'ordre incontournable au vu des urgences environnementales. Elle nécessite la mise en place d'un bilan et d'un plan de transition.

En conséquence, il est primordial de garantir que les entreprises mettent en oeuvre leurs obligations en matière de Beges et adoptent un plan de transition à la hauteur des objectifs fixés. Il y va de la pérennité des activités économiques, et donc des emplois et des compétences. Dans la pratique, le dialogue social est le levier le plus efficace pour construire et suivre une trajectoire de décarbonation adaptée aux réalités

L'unique critère parfois mentionné est l'impact carbone, mais les conséquences sur la biodiversité et la santé, tout aussi essentielles, ne sont pas prises en compte. Dans un contexte de raréfaction des ressources et de multiplication des effets sur la santé humaine et sur la biodiversité, il nous semble nécessaire que ce texte

Le règlement européen Taxonomie met en place une classification des activités en utilisant des critères scientifiques, afin d'aider les investisseurs à identifier les activités durables. Il s'appuie sur six objectifs environnementaux- atténuation et adaptation climatiques, biodiversité, pollution, eau et économie circulaire -et concerne les entreprises de plus de 500 salariés.

pour l'inclure. Dans un contexte où les technologies évoluent rapidement, il nous semble plus pertinent de conserver de la latitude et d'ajuster la liste des industries vertes par voie réglementaire, en fonction des différents aspects abordés par ce texte.

épargne. Nous savons en effet que des fonds éthiques, dont certains sont labellisés par l'État, financent aussi l'industrie pétrolière. Quant au label, il exclut le nucléaire, qui est pourtant une énergie décarbonée.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à mettre l'intitulé du projet de loi en adéquation avec son contenu- c'est la moindre des choses

Dans un contexte de raréfaction des ressources et d'accentuation des répercussions sur la santé humaine et sur la biodiversité qu'emportent les projets industriels, il est nécessaire que ce projet de loi définisse un cadre propice à une politique de réindustrialisation à la hauteur des enjeux sociaux,

Il me semble que tel est l'enjeu premier de toute politique publique en faveur de la réindustrialisation de notre pays. Cet amendement vise ainsi à inscrire ces objectifs essentiels, en complément des objectifs de lutte contre le changement climatique, de développement de l'exploitation des énergies renouvelables

à la lutte contre le changement climatique, au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, à la pollution, à la biodiversité, etc. Le rôle du Sraddet est justement d'articuler et de concilier l'ensemble de ces éléments afin de déployer un aménagement du territoire régional respectueux de ces différents impératifs.

émet donc un avis favorable

elle ne s'inscrit pas non plus dans les trajectoires que le pays s'est fixées, qu'il s'agisse de neutralité carbone, de planification écologique, d'économie circulaire, de sobriété foncière ou encore de biodiversité. Peut-être plus grave encore, aucune référence n'est faite à l'économie qui se met en place

La performance globale des chaînes de valeur ou des parties de chaînes de valeur situées sur le territoire français s'en trouvera ainsi confortée, dans l'intérêt général national. Consolider

du code général des collectivités territoriales, qui ne fait que mentionner les catégories d'objectifs que doit fixer le Sraddet, n'a pas vocation à orienter la politique menée par les régions sur le fond. Pour autant,

explication de vote. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis quelque peu étonné de la manière dont les amendements très précis et détaillés de mon collègue Franck Montaugé sont balayés.

Mme Vanina Paoli-Gagin. En l'état actuel du droit, les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation n'intègrent ni l'occupation des sols ni l'implantation des sites industriels. Or le développement des dynamiques industrielles, avec les flux logistiques qu'elles impliquent, gagnerait à être élaboré au niveau régional. Cela permettrait, d'une part, d'opérer la péréquation des surfaces, dans l'objectif du ZAN, à une échelle plus pertinente, d'autre part, d'intégrer une dimension foncière et logistique dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, en lien avec le développement des transports et l'exercice de la compétence économique. Cet amendement vise donc à renforcer le volet industriel et logistique du Sraddet, en complément de la modification apportée par l'article 1 du présent projet de loi. Il s'agit de renforcer la cohérence des schémas régionaux afin de faciliter la mise en oeuvre de stratégies territoriales cohérentes. Quel est l'avis de

lors de la création des Sraddet, qui limitait les dispositions relevant du domaine législatif aux seuls éléments essentiels des documents sectoriels auxquels le Sraddet s'est substitué, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir, pour chacun des objectifs du schéma, ce qu'il recouvre, ce dont il doit tenir compte et la manière dont il est déterminé. Pour ces raisons,

La réindustrialisation ne se fera pas sans prendre en compte les petites et moyennes industries implantées dans les territoires, leur structuration et leur consolidation. C'est pourquoi nous proposons d'inscrire ces politiques publiques parmi les objectifs et les règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Au travers Solidarité et Territoires souhaite donc optimiser l'intégration de cet enjeu stratégique au sein de la planification régionale. l'avis de la commission ? Mon cher collègue, je vous rejoins quant à la nécessité, pour les régions, de dialoguer avec les collectivités locales pour la fixation des objectifs de développement industriel, afin de substituer à une logique purement descendante une logique de coconstruction. Mais le rapport de prise en compte, mentionné à l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, que vous souhaitez modifier, est un lien juridique. Le Sraddet peut prendre en compte des documents de rang supérieur- stratégies nationales, plans nationaux, etc.

L'association des conseils départementaux à l'élaboration du projet de Sraddet sur les aspects industriels semble, à ce titre, prendre tout son sens. Celle-ci permettra à l'ensemble des collectivités territoriales d'agir de concert afin de favoriser et de faciliter le développement industriel de leurs territoires.

L'article 1 du projet de loi élargit le champ du Sraddet à l'objectif de développement des activités industrielles. En raison des nouveaux enjeux socio-économiques qu'emporte le développement de l'industrie verte sur leur territoire, les départements demandent à être également consultés

Je suis bien sûr tout à fait favorable à cette mesure : c'est en réunissant l'ensemble des parties prenantes- État, collectivités locales, porteurs de projet, aménageurs, etc. -que l'on accélérera

telle utilisation des voies fluviales contribue à la décarbonation du secteur du transport. Le Gouvernement souhaite rendre la France plus attractive pour les industries vertes, et le secteur du recyclage en fait pleinement partie. L'industrie du recyclage se modernise et investit pour s'adapter aux nouveaux gisements de déchets à recycler et pour améliorer ses technologies. Ces investissements sont lourds, de l'ordre de plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions d'euros pour chaque installation. Ainsi, le secteur du recyclage a investi 547 millions d'euros en 2021. Or, à l'heure actuelle, les terrains des zones portuaires sont affectés aux entreprises pour des durées limitées, par le biais d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Si ces autorisations peuvent aller jusqu'à soixante-dix ans, les durées constatées excèdent rarement vingt ans. Elles peuvent constituer un frein réel à l'investissement dans le cadre du développement des activités, puisque les zones portuaires lancent systématiquement une procédure de mise en concurrence dès que la période définie dans l'autorisation arrive à son terme. Afin que les entreprises de recyclage puissent continuer à se développer pour répondre aux défis défis de l'économie circulaire et de la transition écologique, il est nécessaire de sécuriser leurs investissements dans les zones portuaires. Cet amendement vise à prolonger la durée de l'autorisation et à l'aligner sur celle de l'amortissement, en cas de nouvel investissement durant la période définie par l'autorisation. Par ailleurs, cette disposition,

vous proposez de proroger la durée de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public jusqu'à la fin de l'amortissement des investissements effectués dans le cadre de la transition écologique. Lorsqu'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est accordée en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis », 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques. En outre, aux termes de l'alinéa 4 de cet article, la procédure de sélection permettant la mise en concurrence n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une simple prolongation d'une autorisation existante. autorisation existante. Dans le cas d'une exploitation économique, il est simplement précisé que cette prolongation ne peut excéder la durée nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements consentis.

Qu'entend-on par industrie verte ? Quelles sont les filières industrielles à développer prioritairement pour être dans la course du monde économique, social et environnemental souhaitable de demain ?

définie aux échelons national, régional et intercommunal, de manière coordonnée avec les collectivités concernées et les représentants des acteurs économiques. Il rappelle que la notion d'industrie verte ne peut se limiter à la décarbonation et qu'elle recouvre au minimum les industries et les activités contribuant à la neutralité carbone, sans porter atteinte à la biodiversité, aux ressources en eau et à la santé humaine. Notre amendement vise à poser les bases d'une stratégie nationale concertée Industrie verte, afin de disposer d'un socle partagé et d'une trajectoire commune permettant ainsi de mieux appréhender les enjeux de planification industrielle à l'aune des défis économiques, sociaux et environnementaux que nous devons relever et qui feront la France de demain. Quel est l'avis de la

Tous les acteurs publics et privés pertinents y seraient associés, notamment les collectivités, et elle s'appuierait sur les travaux menés par le Conseil national de l'industrie, le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, tout le monde n'a pas été associé à la préparation de ce projet de loi et, plus largement, au programme gouvernemental Industrie verte. Il est donc souhaitable de donner une cohérence aux actions de l'État, des collectivités et de l'ensemble des acteurs en matière d'industrie verte. La commission partage cet objectif d'élaboration d'une stratégie nationale Industrie verte. Aussi émet-elle un avis favorable

mais, à mon sens, celle-ci existe déjà. Il s'agit de la planification écologique que nous sommes en train de finaliser après un an de travail et qui nous permettra de décarboner l'ensemble des secteurs industriels de la France.

l'article 1 , que vous avez adopté en commission et qui modifie les missions statutaires dévolues aux établissements publics fonciers locaux (EPFL), afin qu'ils participent au développement industriel des territoires et à la renaturation en ciblant leur action sur les friches. Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans la loi que les établissements publics fonciers peuvent participer au développement industriel des territoires et à la renaturation.

pour favoriser la limitation de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Les objectifs fixés aux collectivités en matière de sobriété foncière portent sur une réduction de l'artificialisation nette des sols, c'est-à-dire sur le solde entre artificialisation et renaturation. L'intention est donc déjà satisfaite.

qui couvrent pourtant l'essentiel du territoire national et dont les missions sont définies de façon cohérente avec celles des EPF locaux. L'article 1 ainsi voté introduit une forme d'incohérence entre les missions

Monsieur le ministre, vous souhaitez supprimer la précision introduite en commission, selon laquelle les EPFL pourraient acquérir du foncier à des fins d'implantations industrielles, ce qu'ils nous ont déclaré avoir plus de difficultés à réaliser,

pour donner plus de visibilité à certains secteurs et sécuriser les porteurs de projet et les collectivités en matière de déclaration de projet. Pour nous aussi, il s'agit de faire savoir aux EPFL qu'ils sont légitimes

au nom de l'accélération et de la simplification de la mise en oeuvre des projets industriels. Je le rappelle, cet article remplace l'enquête publique par un dispositif de participation spécifique

complexifie le droit et met à mal l'effectivité de la participation du public pour évaluer les impacts d'un projet. Il semble en effet impératif de prévoir au moins un mois de consultation du public après

la procédure d'instruction des autorisations environnementales. Il cherche ainsi à renforcer l'attractivité industrielle de notre pays. La nouvelle procédure de consultation permet également de répondre aux demandes de participation de nos concitoyens. Organisée plus tôt qu'aujourd'hui, cette

sont de nature à assurer une participation effective du public. À son sens, elles ne soulèvent pas de difficultés au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article 6 de la directive 2011/92/UE, dès lors qu'elles s'attachent à concilier une association précoce du public au processus de décision et la possibilité, pour le public, d'être éclairé par les avis remis avant de produire ses propres observations, en allongeant le délai de consultation à trois mois. Néanmoins, le caractère raisonnable du délai de trois mois fixé pour le déroulement simultané des phases d'examen et de consultation paraît peu opérant si l'on se place du point de vue du pétitionnaire. En effet, les observations et propositions parvenues pendant la phase de consultation devront être prises en considération par le maître d'ouvrage, qui pourra ainsi être tenu d'adapter son projet. Les réponses et propositions de modifications qui devront être apportées par le pétitionnaire auront toute leur importance, car elles seront réputées faire partie du dossier de demande. Or la prise en compte au fil de l'eau des observations du public et avis des autorités par le pétitionnaire pour apporter des réponses et précisions

Cette mesure, qui bénéficie à tous les acteurs, permet de prévenir des atteintes illégales à l'environnement : la simplification ne doit pas être menée au détriment des garanties contentieuses. en vigueur, le juge ne pourrait plus suspendre un projet contesté soumis à un référé-suspension. C'est là une porte ouverte aux atteintes illégales à l'environnement. Ainsi, un projet industriel pourrait être lancé, puis déclaré illégal quelques mois plus tard, mais le mal serait fait : les travaux auraient été effectivement engagés. La suspension automatique a précisément ce rôle : empêcher l'ouverture de travaux sérieusement susceptibles d'être illégaux.

les délais d'installation. Cela étant, les citoyens peuvent toujours demander au juge des référés de suspendre la décision d'autorisation environnementale. De même, dans sa décision, le juge administratif peut toujours prendre en compte les conclusions motivées du commissaire enquêteur. Pour ces raisons, la commission émet

précise bien que le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise, sans que la participation du public mentionnée à l'article L. 123-1-1 ait eu lieu, alors qu'elle était requise. Nous nous contentons de transférer la